Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits des missions

je commencerai par évoquer la mission « Gestion des finances publiques ». Dotée de plus de 10 milliards d'euros, cette mission porte les crédits des deux grandes administrations de réseau de Bercy que sont la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Permettez-moi d'abord un premier constat : si l'heure ne semble plus être à la maîtrise de nos dépenses publiques, la mission « Gestion des finances publiques » continue de montrer l'exemple ses crédits sont en baisse, tout comme ses dépenses de personnel. Ce n'est pas rien pour une mission qui porte près de 117 000 équivalents temps plein (ETP). Les administrations de la mission ont été particulièrement mobilisées durant la crise sanitaire. Je pense notamment à la DGFiP. La direction a dû continuer d'exercer ses activités traditionnelles essentielles, tout en remplissant de nouvelles missions. On lui a ainsi confié la gestion du fonds de solidarité et elle a effectué un travail de veille sur les entreprises, les collectivités et les hôpitaux.

Pour les douanes, le premier des enjeux est bien sûr le Brexit, cette échéance étant de plus en plus proche. Paradoxalement, et je pense qu'on ne le dira pas souvent dans cet hémicycle, la crise sanitaire et économique devrait avoir un effet positif. Elle a en effet conduit à une chute brutale du volume des échanges et des trafics, aériens comme routiers. Ces moindres échanges devraient faciliter la période de transition. Pour la DGFiP, et je pense que cela nous tient tous très à coeur, le grand enjeu reste la réorganisation de son réseau. On nous promet un réseau de 1 200 conseillers aux décideurs locaux, mais à peine 5 % d'entre eux sont déjà en place. On nous promet une augmentation de 30 % du nombre de points de contact pour les usagers, mais dans quelles conditions ? Grâce à un bus présent une demi-journée par semaine ? Est-ce vraiment là ce que nos concitoyens appellent de leurs voeux quand ils parlent de la proximité des services publics ? Je n'en suis pas sûr On nous promet enfin la délocalisation de certains services. C'est vrai, mais pas avant 2023 ou 2024 pour l'essentiel, et tous n'auront pas vocation à accueillir du public. Je rappelle par ailleurs que les collectivités sont fortement mises à contribution pour accueillir ces services, ainsi que les maisons France Services. J'espère que le Gouvernement saura nous rassurer sur ses promesses. Le troisième enjeu concerne la gestion des ressources humaines, essentielle quand on parle de 117 000 emplois. Les transformations en cours appellent à la révision des règles de mobilité ou de rémunération. Enfin, le contrôle fiscal Le Gouvernement aura beau jeu de nous présenter des résultats record pour 2019, n'oublions pas qu'ils viennent après une baisse ininterrompue de trois ans ! Ce n'est pas peu dire pourtant que le commerce électronique, qui explose aujourd'hui, est porteur d'un risque de fraude décuplé.

le déploiement du forfait mobilités durables dans la fonction publique d'État ; des revalorisations indemnitaires, décidées lors du rendez-vous salarial de la fonction publique il y a trois mois. Or, et nous le regrettons vivement, la ventilation des crédits entre ces trois mesures n'est pas précisée. Pour nous, c'est un manque de transparence alors que cette dotation atteint un montant exceptionnellement élevé : près de 200 millions d'euros en 2021, contre 26 millions d'euros seulement en 2020. Lors de l'examen des crédits de la mission en commission, nous espérions que le Gouvernement procéderait à cette répartition d'ici à la séance, mais tel n'a pas été le cas. Pour conclure, il me revient de vous faire part de la position de la commission sur ces deux missions : nous vous proposons d'adopter leurs crédits. Pour la mission « Gestion des finances publiques », il s'agit de signifier notre soutien vigilant aux processus de rationalisation engagés. La parole

On nous parle également en parallèle de dématérialisation des services publics, mais dans quelles conditions peut-elle se faire ? Certes, la numérisation doit permettre aux administrations d'être plus efficaces.

Je vais maintenant vous présenter le compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ». Globalement, ce compte présente peu de changements.

qu'on a confié une mission à un expert sur la revalorisation des biens inutiles à l'État. On attend toujours ses propositions et ses traductions concrètes, alors que cela fait des années que notre commission des finances

servir de vecteur budgétaire. Pourtant, ses recettes et ses dépenses connaissent une baisse tendancielle. Dans ces conditions, on voit mal comment on parviendra à financer tous les besoins d'un parc immobilier dégradé. Le CAS ne suffira pas à porter les grands projets de l'État dans le domaine immobilier.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission « Régimes sociaux et de retraite » couvre tout ou partie des besoins de financement de dix régimes spéciaux de retraite déficitaires du fait de leur déséquilibre démographique rendant obligatoire la contribution de l'État solidaire. Pour Pour 2021 cette contribution s'élèvera à 6,153 milliards d'euros, en baisse de 74,2 millions par rapport à 2020. Les deux tiers sont pour la SNCF, la RATP

Je rappelle que le projet de loi instituant un système universel de retraite a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 3 mars 2020, avant d'être mis en sommeil par le Président de la République. Le 15 juillet 2020, le Premier ministre Jean Castex a toutefois rappelé l'objectif de « créer un système universel de retraite qui implique clairement la disparition à terme des régimes spéciaux tout en prenant pleinement en considération la situation des bénéficiaires actuels de ces régimes Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer le contenu et la lisibilité de la réforme la reprise d'une concertation. Les parlementaires seront-ils associés à cette étape ? Je ne dispose d'aucun élément sur ce point, pas plus que sur l'équité ou la soutenabilité de la réforme. Hors réforme et pour 2021, je précise que les crises sanitaires en cours sont susceptibles d'avoir des effets sur les comptes de la mission. Une surmortalité parmi les pensionnés des régimes des mines a été observée dans les régions Île-de-France et Grand Est.

mais on l'attend toujours, ce qui fragilise d'autant le financement du régime. Je dirai maintenant un mot sur la contribution solidaire et nécessaire de l'État à l'ensemble de ces régimes spéciaux déficitaires.

Pour la SNCF et la RATP, le coût supporté par l'État s'élèverait à 970 millions d'euros annuels, selon la Cour des comptes. Une réforme sur ce point serait la bienvenue, et c'est en grande partie l'objet de celle qui est projetée. « Pensions » retrace les opérations relatives aux pensions civiles et militaires de retraite et d'invalidité des agents de l'État : 60,2 milliards d'euros sont prévus pour 2021, dont 56,7 milliards d'euros pour les seules pensions civiles et militaires 1,94 milliard d'euros pour les ouvriers des établissements industriels de l'État ; 1,54 milliard d'euros pour les pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.

qui est toujours supérieure aux dépenses. Pour mémoire, le taux des cotisations patronales est de 74 % pour les civils et de 126 % pour les militaires. Ces taux sont appliqués à la masse salariale de chaque ministère, puis imputés sur les programmes des ministères employeurs. L'excédent prévisionnel est de 759 millions pour 2021. Le solde cumulé du CAS « Pensions » atteindrait donc 9,9 milliards d'euros Notez la substantielle contribution du CAS « Pensions » à l'équilibre général du système de retraite puisque le déficit de la branche vieillesse ne cesse de se creuser. Le solde cumulé du CAS « Pensions » devrait continuer de croître jusqu'en 2027, puis devenir légèrement négatif jusqu'en 2063, fin de la génération du papy-boom. Notons cependant que l'État emploie de plus en plus de contractuels, qui alimentent non pas le CAS « Pensions », mais la CNAV, ce qui se traduit par une baisse de recettes immédiate, mais par des économies à long terme, car les pensions seront moins nombreuses. Au terme de ces observations, je vous propose d'adopter l'ensemble des crédits de la mission, soit 66,4 milliards d'euros.

le rappelle, le solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse atteindra 11,4 milliards d'euros l'an prochain.

par la subvention d'équilibre apportée par cette mission. Aussi, si des déséquilibres démographiques sont compensés au sein de notre système par répartition, il n'apparaît pas légitime de financer par la solidarité nationale des avantages persistants en termes de conditions de départ à la retraite. La commission a donc renouvelé sa réserve sur ces crédits. La commission a constaté également que, pour la première fois, le compte d'affectation spéciale portera

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, je tiens à saluer l'engagement et la réactivité des 5,56 millions d'agents publics qui sont en première ligne pour assurer la continuité du service au public face à l'épidémie que nous connaissons, et ce dans les trois fonctions publiques. Le projet de loi de finances pour 2021 acte définitivement le renoncement du Gouvernement à réduire les effectifs de l'État, comme il s'était engagé à le faire à hauteur de 50 000 emplois. En effet, seulement 147 postes seront supprimés dans la fonction publique de l'État. Au total, un peu plus de 2 000 équivalents temps plein ont été supprimés depuis 2018, bien loin des efforts nécessaires pour compenser la création de plus de 26 000 ETP entre 2013 et 2017. le programme 148, « Fonction publique », finance les actions interministérielles en matière de formation, d'action sociale et de gestion des ressources humaines. Il s'établit à 224,37 millions d'euros en crédits de paiement, soit une hausse notable de 6,87 %. En termes de formation, je relève l'effort louable pour développer les classes préparatoires intégrées (CPI). Il en existe aujourd'hui 27, qui accueillent 714 élèves. Le Gouvernement prévoit de créer 1 000 places, pour un coût de 7 millions d'euros, de doubler le montant de l'allocation pour la diversité, qui passerait de 2 000 à 4 000 euros par élève. Je regrette toutefois que le modèle des CPI ne soit pas étendu à la fonction publique territoriale, dans laquelle il conviendrait aussi d'encourager la diversité des profils. En ce qui concerne l'action sociale, le budget interministériel augmente de 5,3 millions d'euros afin de financer les engagements pris par le Gouvernement lors du rendez-vous salarial de juillet 2020. Cependant, une fois encore, je souhaite attirer votre attention sur l'apprentissage dans la fonction publique. L'État s'était engagé à employer 10 000 apprentis à la rentrée 2016. Quatre ans plus tard, cet objectif n'est toujours pas atteint, loin de là. Le nombre d'apprentis a même baissé de 25 % en deux ans : on en compte à peine plus de 7 000 dans les services de l'État en 2019. Si les collectivités territoriales font figure de bons élèves, avec près de 60 % des contrats conclus, l'État, lui, a pris du retard, alors même que la France n'a jamais compté autant d'apprentis. 491 000 contrats étaient en cours en 2019. Comme l'année dernière, je tiens à pointer le manque de coordination entre les ministères. En l'absence de cadrage national, chaque ministère doit négocier les conditions de prise en charge de ses apprentis avec les centres de formation d'apprentis (CFA), ce qui constitue une perte d'efficacité. Je regrette la suppression de la dotation interministérielle pour le financement de l'apprentissage. Afin d'inciter les ministères à recruter des apprentis, je vous proposerai un amendement visant à recréer cette dotation de 15 millions d'euros, à l'instar de ce que prévoyaient les lois de finances entre 2016 et 2018.

Tout d'abord, je suis au regret de rappeler que cette mission connaît depuis plusieurs années des baisses de crédits constantes et inquiétantes. Ces réductions drastiques placent la DGFiP parmi les administrations ayant fait l'objet du plus grand nombre de suppressions de postes ces dix dernières années.

Cette suppression peut paraître anachronique au regard des enjeux et défis qu'auront à relever les services de la DGFiP l'année prochaine, les principaux étant le contrôle et le recouvrement de l'impôt. Avec ces baisses de crédits, l'État organise son impuissance dans la lutte contre la fraude fiscale, et ce sont bien sûr les petits contribuables, respectueux des lois, qui paient la facture

tête des premiers perdants figurent les États-Unis, l'Allemagne et, malheureusement, la France. Nous sommes médaillés de bronze de l'évasion fiscale alors que nous devrions avoir un percepteur qui vise la médaille d'or. Force est de constater que vos coupes budgétaires ne nous permettent pas d'espérer de figurer sur le podium en matière de recouvrement fiscal des fraudeurs. Vos coupes budgétaires ont aussi des effets sur les défis que notre pays doit relever. Je rappelle que ce sont les personnels de la DGFiP qui doivent piloter la mise en place des fonds de soutien intégrés dans le plan de relance. Chacun appréciera la duplicité qui vous anime sur ce sujet. Vous claironnez dans les médias que vous allez redynamiser le pays avec le plan de relance alors même que vous ne mettez pas assez de moyens matériels pour en assurer le suivi. À la suppression de ces 1 800 ETP s'ajoute la fermeture programmée de près de 1 000 trésoreries au cours de l'année qui arrive. Ces trésoreries permettent aux usagers, aux petites entreprises, aux collectivités territoriales d'obtenir de précieux conseils fiscaux. La dématérialisation ne résoudra pas tout. Il suffit d'écouter Bruno Parent, ancien directeur général de la DGFiP pour s'en convaincre. Il déclarait en 2016, lors d'une audition à l'Assemblée nationale : « La dématérialisation ne peut se substituer à l'accueil de public pour qui la fracture numérique est une réalité ». La fracture numérique est un concept sûrement très vague pour la « start-up nation », mais elle est pourtant bien réelle dans nos territoires. En réduisant encore les crédits de cette mission, vous privez la France des moyens de lutter contre l'évasion fiscale tout en organisant l'attrition de nos finances publiques. De plus, vous sacrifiez le service et l'assistance des trésoreries dans nos territoires, en prétendant qu'ils trouveront leur salut dans la dématérialisation ou dans les maisons France Services. Nous ne partageons pas cette vision. En conséquence, nous ne voterons pas les crédits de cette mission.

attiré mon attention. Le premier concerne le financement du forfait mobilités durables, qui est une aide versée par l'employeur pour financer des trajets domicile-travail moins polluants.

Malheureusement, celui-ci est aujourd'hui toujours facultatif. L'effectivité des mesures prises par le Gouvernement et sa volonté de reprendre sans filtre les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat pour les soumettre à un vote montrent encore une fois leurs limites.

les 400 euros par an, la mesure ne profite pas aux salariés qui prennent un abonnement pour les transports en commun. Le deuxième point est relatif au financement de la prime de fidélisation destinée aux fonctionnaires de la Seine-Saint-Denis.

se remarque encore dans la mission « Gestion des finances publiques ». La volonté du Gouvernement de s'entêter dans une politique de dématérialisation et de concentration des centres d'impôts dans les zones urbaines est aussi un signe de cet éloignement grandissant.

L'accès physique au service public pour les collectivités comme pour les particuliers disparaît petit à petit. Dans le même temps, le déploiement et le fonctionnement du réseau numérique sont très variables. Cela pénalise les zones rurales, qui sont les premières à voir le service public s'éloigner des citoyens.

les missions « Gestion des finances publiques » et « Transformation et fonction publiques » regroupent les crédits qui participent activement à la transformation de l'action publique, s'inscrivant en cela dans la dynamique engagée voilà trois ans. et droits indirects (DGDDI) devront poursuivre leurs efforts pour combler leur retard technologique et numérique et repenser leurs métiers comme leurs procédures. La baisse des crédits constatée en 2021 s'explique dès lors presque exclusivement par la baisse des dépenses de personnel. La mission « Transformation et fonction publiques » retrace les crédits interministériels destinés à soutenir directement la transformation publique. Les programmes de cette mission, dont les crédits augmentent de 10,7 % par rapport à 2020, constituent la traduction opérationnelle et budgétaire d'Action Publique 2022. Nous nous réjouissons ainsi de voir les crédits du programme 148, consacré à la formation des fonctionnaires, à l'action sociale interministérielle et à l'appui et à l'innovation des ressources humaines, augmenter de 3,5 %. mentionner la hausse des dépenses informatiques, du montant des allocations pour la diversité dans la fonction publique et la bonne mise en oeuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations. Lors de l'examen de la mission à l'Assemblée nationale, l'adoption d'un amendement du Gouvernement a permis d'augmenter de 1 000 le nombre de places en classes préparatoires intégrées. Avec le doublement de l'allocation diversité, c'est un geste de plus en faveur du renforcement de l'égalité des chances dans dans l'accès à la fonction publique. Les crédits de paiement de cette mission se caractérisent néanmoins par une sous-consommation importante, notamment s'agissant de la rénovation des cités administratives. Nous attendons que le ministre lève les inquiétudes qui ne manqueront pas de s'exprimer sur nos travées. Les recettes prévisionnelles du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » diminuent légèrement, de 2,63 %, en raison des mauvaises perspectives économiques. Notons cependant que le volet immobilier du plan de relance prévoit une allocation sans précédent de 3,7 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments de l'État. Le programme 551 de la mission « Crédits non répartis » fait l'objet d'une demande de crédits, pour la quatrième année consécutive. Elle s'élève cette année à 198,5 millions d'euros, contre seulement 16 millions d'euros en 2020. Elle permettra de financer le forfait mobilités durables, la prime de fidélisation en Seine-Saint-Denis et diverses mesures annoncées dans le cadre du rendez-vous salarial du mois de juillet 2020. La mission « Régimes sociaux et de retraite » voit ses crédits diminuer de 1,9 % cette année, pour atteindre 6,15 milliards d'euros. Toutefois, si l'on considère les besoins de financement observés en 2020,

Pensions » enregistreront en 2021 une hausse de 1,03 % par rapport à 2020. Si le solde cumulé continue d'augmenter dans le PLF pour 2021, l'excédent dégagé connaît une diminution de 46,37 %, en raison notamment du gel du gel du point d'indice et du vieillissement de la population. Le groupe RDPI vous invite à adopter les crédits de ces différentes missions, qui, à mon avis, font l'objet d'un large consensus au sein de notre assemblée. La parole

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, je regrette de devoir encore une fois évoquer en quelques minutes les enjeux de quatre missions et de deux comptes spéciaux. J'irai donc droit au but, comme on dit à Marseille Pour commencer, je m'attarderai particulièrement sur la mission « Gestion des finances publiques », qui constitue la principale mission du pôle économique et financier de l'État. L'administration fiscale et les douanes représentent 91 % des crédits de cette dernière. Je salue la simplification de l'intitulé de cette mission. Les remarques que nous avions formulées l'an dernier semblent avoir été entendues sur ce point. Gageons que l'amélioration de la lisibilité et de l'intelligibilité continuera. Je me félicite également

Je salue ainsi l'ambition du Gouvernement de déconcentrer et de « démétropoliser » ces administrations, qui ont trop d'effectifs en administration centrale, et pas assez sur le terrain, à proximité des usagers, des élus locaux et, bien trop souvent, des problèmes qu'elles ont à traiter. Cela va dans le bon sens, d'autant que la crise sanitaire nous rappelle la nécessité d'accélérer la déconcentration des services centraux pour mieux répondre aux besoins des populations. Pour autant, ne tombons pas dans le piège d'une décentralisation en trompe-l'oeil ces réorganisations territoriales doivent se faire au minimum en concertation avec les acteurs de l'échelon local, afin de mieux répondre aux enjeux spécifiques de chaque territoire. Nous ne devons pas condamner inutilement des antennes locales de l'administration fiscale. Par ailleurs, nous restons sensibles au devenir de l'administration des douanes, qui connaît d'importantes remises en question de ses missions. Dans tous les cas, nous attendons beaucoup du futur projet de loi « 3D » pour rationaliser et optimiser la décision publique locale, entre État et collectivités. La mission « Transformation et fonction publiques » voit son périmètre modifié par l'intégration du programme 148, « Fonction publique ». Je constate une annulation de 75 % des crédits de paiement en raison des retards accumulés sur la contractualisation des projets financés par les fonds de cette mission. À l'instar des rapporteurs, je regrette que le Parlement ne dispose pas d'indicateurs plus efficaces permettant de suivre l'évolution des projets, alors qu'une de nos principales missions est le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre de la loi ... quand nous en avons le temps Je note ensuite une hausse marquée des « crédits non répartis », répondant ainsi aux dépenses imprévisibles liées à la crise sanitaire. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles La hausse du budget des pensions des agents publics devrait continuer de ralentir. J'attire votre attention sur le fait que la programmation de ces crédits se fonde sur des hypothèses dont la concrétisation échappe en partie au pilotage des gestionnaires, la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques n'ayant pas été actualisée. Je ne puis que m'interroger sur l'ampleur de l'écart entre la prévision et la réalisation de ce budget, qui apparaît ainsi assez incertain. Je terminerai en évoquant le compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ». Il me semble plus que nécessaire de lancer une réflexion commune sur le devenir du parc immobilier de l'État. Au-delà des problématiques habituelles, comme le manque de politique unifiée, la maîtrise des coûts ou la rénovation énergétique, la crise sanitaire a largement modifié nos pratiques en généralisant le recours au télétravail.

La question mérite d'être posée au vu du nombre effarant de suppressions d'emplois et de la part principale que cela prend dans ce budget. La prévision de suppression de postes en 2021 est conforme aux annonces de 2020. Ce sont ainsi 4 900 postes qui disparaîtront d'ici à la fin du quinquennat. Les rapporteurs spéciaux notent également que la DGFiP contribuerait pour un tiers à l'objectif révisé de 15 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'État fixé par le Gouvernement. est donc de loin celle qui contribue le plus à la « rationalisation » de la masse salariale publique. Lors de leurs auditions, les rapporteurs spéciaux ont demandé aux responsables des trois programmes de la mission jusqu'à quand et à quel niveau ils estimaient que ces réductions d'effectifs pouvaient se poursuivre. Selon eux, il arrivera en effet un « palier où les gains de productivité ne suffiront plus à compenser la réduction des effectifs ». Ce processus continu de réduction des effectifs trouve toujours une justification différente. tantôt au nom d'une rationalisation de la présence territoriale, tantôt au nom de la modernisation des outils, quand ce n'est pas au nom de la dématérialisation des procédures fiscales et du recours à l'intelligence artificielle. Mais enfin, mes chers collègues, comment tolérer une baisse de 1,56 % du budget du programme chargé du recouvrement de l'impôt d'État et du secteur public local ? Cela représente une diminution de 123 millions d'euros de dépenses de personnel ! Nous savons pourtant bien que les grandes entreprises utilisent des montages toujours plus complexes pour échapper à leurs obligations fiscales, que les géants du numérique, mis en cause ces temps-ci, refusent de s'acquitter de leur impôt, préférant le contentieux, puis un arrangement avec l'administration, et que les niches fiscales rendent toujours plus difficile de définir le juste montant. Pour rappel, une dépense fiscale sur deux a fait l'objet d'un chiffrage sur la base d'un « ordre de grandeur » ou, pire encore, n'a pas été chiffrée du tout ! Nous ne pouvons nous satisfaire que plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales de l'État comme des collectivités locales soient perdus au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements faute d'avoir pu engager les voies et moyens nécessaires à leur recouvrement. L'administration fiscale, par manque de moyens, s'incline devant l'ingénierie des fraudeurs et la malice des tricheurs. Elle renonce parfois, de guerre lasse. J'en veux pour preuve deux indicateurs. seuls 12 % des dossiers répressifs ont été transmis au parquet en 2020. C'est la part des dossiers transmis à l'autorité judicaire sur la base de la lutte contre la fraude fiscale et l'escroquerie. C'est, bien entendu, largement insuffisant. Il est probable que ces signalements seraient plus nombreux si les moyens d'investigation étaient accrus. D'autre part, 67 % des créances issues du contrôle fiscal externe ou sur pièces sont réellement encaissées, à l'exclusion des créances sur lesquelles les comptables ne peuvent pas agir. Un tiers des contrôles fiscaux font donc l'objet d'une mesure de recouvrement qui n'aura jamais lieu l'impuissance de l'administration fiscale, toujours l'impuissance ... Cette impuissance se manifeste également lorsque la France se contente d'un « règlement d'ensemble » de 523 millions d'euros avec Google, renonçant ainsi au moins au double du montant qu'espérait la DGFiP. À son bon vouloir, Google a décidé de « transiger » avec la justice et l'administration fiscale. Cette perte de ressources entérine également une convention fiscale dérogatoire dont nous ne connaissons pas les termes. Qu'est-ce qui a été négocié ? Cette affaire avait été qualifiée d'« hors norme » par un représentant du parquet national financier. Il est impératif que, en face, les moyens consacrés à la lutte contre à la fraude et l'évasion fiscale soient également « hors norme » ou, au moins, à la hauteur. Le coût de collecte des recettes douanières et fiscales n'est que de 73 centimes pour 100 euros.

le 29 octobre dernier, la ministre du travail déclarait que le télétravail était, non pas « une option », mais bien une « obligation » qui serait « inscrite dans le nouveau protocole national en entreprise » et que « le temps de travail effectué en télétravail » était « porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer leurs tâches à distance

a mis en lumière la forte dépendance des modes de travail actuels aux technologies numériques. Les investissements contraints des années antérieures ont eu de fortes conséquences sur un taux d'équipement limité des agents en matériel de bureautique portable

à la fin de l'année 2020. On comprend bien que le télétravail était compliqué ... Dans un autre ministère, alors que le télétravail était interdit

Cela me semble contrevenir au décret du 5 mai 2020, qui est venu actualiser le décret de 2016 sur le télétravail dans la fonction publique. Dans ce même ministère, dont je tairai le nom, les services support refusent catégoriquement d'installer du matériel personnel, une imprimante, sur l'ordinateur portable de l'agent en télétravail : « Absurdistan » ! Au-delà de l'équipement, ce sont aussi les procédures qui doivent être dématérialisées et simplifiées. Certains ici se rappelleront peut-être comme moi avec nostalgie du parapheur qui monte et qui redescend entre les échelons hiérarchiques pour changer une virgule ou un mot. Je me souviens aussi de la complexité de la gestion des courriers parlementaires, avec l'absence d'un fichier partagé entre le cabinet du ministre et l'administration centrale. centrale. Heureusement, au ministère de la transition écologique, la modernisation est « en marche » ! En 2021 sont prévus des travaux relatifs à la mise en cohérence des dispositifs de gestion du courrier, la mise en place du parapheur électronique, la préparation du recours au vote électronique pour les élections professionnelles de 2022 ou encore le développement des libres-services agents et la dématérialisation des actes administratifs dans la gestion des ressources humaines, le déploiement d'un système d'information (SI) d'archivage électronique ou l'interconnexion des premiers SI. Les collectivités territoriales sont vraiment bien en avance

appelle la fraude : plus le système est complexe, plus les fraudeurs peuvent agir facilement. La simplification de notre système fiscal, notamment au regard du nombre de dispositifs dérogatoires, les fameuses « niches fiscales », serait le meilleur moyen de limiter les coûts, d'améliorer l'efficience et de redéployer les agents de la DGFiP vers le contrôle fiscal.

beaucoup plus important que ce qui existe aujourd'hui. La direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) manque d'expertise,

par de l'évasion fiscale à Jersey et au Luxembourg. Il y a tout de même des problèmes sur ces schémas d'optimisation fiscale ! Je sais que le nombre de contrôles et de validations a été augmenté. Mais j'ai tendance à penser que l'inopposabilité de ce type de schémas s'ils n'ont pas fait l'objet d'un accord des services

le réseau conventionnel est extrêmement important. Les enjeux budgétaires sont extrêmement élevés. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les pertes de recettes

le compte n'y est pas, ni dans les modalités de contrôle ni dans la récupération des fonds. La moitié des pays européens utilisent le même logiciel de détection précoce.

et à mesure que le système se développe, les fraudeurs sont de plus en plus malins. Or un fraudeur satisfait est un fraudeur qui revient ... Monsieur le ministre, faites en sorte qu'ils ne reviennent pas

les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite », sur lesquels je m'exprimerai, et du compte d'affectation spéciale « Pensions » sont globalement en baisse de 1,19 %, pour un montant de 6,15 milliards d'euros en 2021.

Ces dépenses seront de plus de 60 milliards d'euros en 2021. C'est la première fois que l'on note une hausse de ce compte d'affectation, à hauteur de 1,03 %.

par rappeler un fait : lors de la dernière réunion du Conseil d'orientation des retraites, il a été clairement établi que notre système de retraite avait retrouvé l'équilibre en 2019, avant la crise sanitaire.

La crise est passée par là, et les déficits actuels sont, à l'évidence, extraordinaires. Faut-il pour autant se précipiter et annoncer qu'il incombera aux seuls salariés de payer la facture,

Quelle curieuse façon de donner confiance en l'avenir aux Français, premières victimes de la crise, en leur promettant pour seul horizon des restrictions et une vieillesse de pauvreté Quelle curieuse façon de promouvoir la cohésion sociale, en disant toujours aux mêmes qu'ils devront payer et toujours aux mêmes qu'ils resteront bien au chaud !

Valéry Giscard d'Estaing disait : « Les Français d'aujourd'hui ont du mal comprendre la société dans laquelle ils vivent. » Ces mots trouvent encore écho dans la période que nous traversons. En effet, beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas toujours les transformations de notre société et appréhendent l'avenir. Pourtant, les Français sont aussi parfaitement conscients que le temps du changement est inévitable, alors que nous faisons face à une crise multiple. L'action publique doit donc impérativement s'inscrire dans cette perspective, et il convient d'évaluer les missions « Gestion des finances publiques » et « Transformation et fonction publiques » au regard de ce contexte si particulier. particulier. La mission « Gestion des finances publiques » contient des changements majeurs dans ce PLF 2021. Elle est particulièrement marquée par la transformation des missions de la direction générale Pour la DGFiP, une réorganisation territoriale se met en place afin de former un « nouveau réseau de proximité », qui se traduit par l'augmentation du nombre de points de contact sur le territoire, la délocalisation des services des métropoles vers les villes moyennes et la création d'un réseau de conseillers auprès des décideurs locaux. Vous connaissez toutefois les craintes exprimées par les élus locaux, qui sont attachés à leurs trésoreries dans leurs territoires. Il est nécessaire de maintenir un accueil physique et téléphonique. La mission « Gestion des finances publiques » marque également un changement fondamental pour la DGDDI, avec le transfert de la gestion du recouvrement des taxes et impositions vers la DGFiP. Si le souhait d'avoir un portail unique à la DGFiP est tout à fait louable, ce changement remet en question les missions essentielles de la douane. J'ai notamment été alerté, dans ma circonscription, Ce transfert des missions pourrait donc être l'occasion de s'interroger sur les missions de la douane dans le futur, à l'heure du Brexit, de l'augmentation du commerce électronique et de la fraude.

Au vu des chiffres, la priorité doit se porter sur la lutte contre la fraude à la TVA, estimée à plusieurs milliards d'euros. Mettons-nous à la place d'un petit commerçant « non essentiel fermé pendant plusieurs mois et qui a vu le commerce numérique s'amplifier, avec des acteurs qui ne respectent pas toujours les règles du jeu. Nous faisons face ici à un enjeu qui entraînera nécessairement une transformation de l'action publique dans ce domaine. J'en viens donc désormais à la mission « Transformation et fonction publiques », qui doit construire l'action publique et l'État de demain. L'action publique de demain doit être celle des territoires et de la proximité. La proximité, c'est remettre la décision au plus proche de nos concitoyens. Les élus locaux ont tous vécu cette crise difficilement, non seulement par la verticalité, mais aussi par une incompréhension des décisions prises à Paris. Il faut déconcentrer au maximum les décisions de l'État et responsabiliser les acteurs locaux. La proximité, c'est aussi l'accessibilité du service public. Avec la démarche France Services, l'État va enfin se réengager dans les territoires et répondre à ce besoin de proximité. Cette accessibilité des services publics se fera également par l'intermédiaire du numérique, qui va transformer en profondeur l'action publique. Certes, le Gouvernement veut s'engager sur la 5G, mais de nombreuses zones de nos territoires ont encore une mauvaise connexion internet. internet. L'action publique de demain doit aussi être facilitatrice avec les différents acteurs, notamment les élus locaux et les collectivités locales. L'État ne doit plus se contenter du contrôle de légalité ; il doit devenir un véritable partenaire pour porter, au côté des collectivités, les projets structurants dans nos territoires. Enfin, la fonction publique de demain est celle qui met en place une réelle stratégie de gestion des ressources humaines. L'État est de moins en moins attractif pour l'ensemble de la fonction publique, particulièrement chez les jeunes. Outre la question des rémunérations, il faut donner des perspectives d'évolution de carrière aux personnes qui font le choix de la fonction publique. En conclusion, les chantiers sont nombreux, mais ils sont primordiaux pour tendre vers un État plus proche, plus efficace, plus juste et plus attractif. Comme le disait Valéry Giscard d'Estaing : « Gouverner, c'est réformer.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est un honneur pour moi de présenter devant vous cette nouvelle mission « Transformation et fonction publiques »,

au sein de la fonction publique redevienne un moteur pour l'ensemble de la société et que nous puissions regagner en attractivité, comme le soulignait M. le sénateur Klinger. Le Président de la République a appelé de ses voeux une petite révolution dans l'accès aux grands concours.

Cette mission budgétaire, comme mon ministère, porte l'ambition de transformer durablement et profondément notre action publique. La crise que nous traversons et la relance que nous devons impulser commandent d'amplifier cette action

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, pour commencer, souligner que les administrations qui portent les crédits évoqués aujourd'hui ont été au premier plan dans la mise en oeuvre des réponses économiques à la crise sanitaire. Je veux saluer leur réactivité et le plein engagement des agents. Je pense notamment à la direction générale des finances publiques, qui a su mettre en oeuvre notre plan de soutien massif à l'économie dans un contexte très dégradé. J'ai toujours plaisir à rappeler qu'il a fallu moins de deux semaines pour mettre sur pied le fonds de solidarité.

et la DGFiP continuent de développer des réponses à destination des entreprises en matière de gestion de la crise. Je pense notamment à la mise en place d'un numéro de téléphone unique pour répondre aux questions des chefs d'entreprise et des indépendants confrontés à des difficultés, et améliorer ainsi le niveau de recours aux aides. aides. Cette réactivité de nos administrations durant la crise sanitaire a confirmé la pertinence et la nécessité des chantiers de transformation numérique et de modernisation des systèmes d'information, en particulier à la DGFiP et à la direction générale des douanes.

garantir aux élus locaux une qualité de conseil en déployant 1 500 conseillers aux décideurs locaux installés au plus près des territoires dans les maisons France Services, dans les implantations de la DGFiP ou encore dans les locaux occupés par les intercommunalités ou les collectivités partenaires C'est également le cas de la réforme du recouvrement fiscal et social, chantier d'ampleur qui vise à rationaliser l'organisation du réseau de recouvrement en valorisant un interlocuteur unique dans chaque sphère pour le recouvrement des prélèvements obligatoires. Nous allons créer un portail unique de recouvrement des créances sociales et fiscales pour faciliter la vie des entreprises. Enfin, la direction générale des douanes se prépare également à faire face à l'augmentation du nombre de déclarations avec la fin de l'exonération pour les envois dits de « valeur négligeable

Les réformes que nous menons depuis trois ans permettent d'importants gains de productivité, et c'est la raison pour laquelle la mission « Gestion des finances publiques » voit ses crédits de paiement diminuer de 1,3 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ce qui traduit les efforts de maîtrise des dépenses et de réorganisation des administrations. Le plafond d'emplois est fixé à 120 043 ETP, soit 1 539 de moins qu'en 2020. C'est aussi le résultat de transformations efficientes de l'administration que je tiens à saluer. Je termine en un mot sur les questions immobilières.

à trouver d'autres moyens de valorisation du patrimoine de l'État, notamment en dynamisant les redevances domaniales et en cherchant des alternatives à la cession. Nous travaillons actuellement à la conclusion de baux de longue durée, qui permettront à l'État de trouver des recettes sans renoncer à la propriété d'éléments patrimoniaux importants. Nous veillons aussi,

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues,

pourront en témoigner -, nous subissons des décisions péremptoires de l'État qui aggravent le processus de désertification. En tant qu'ancien maire et président d'intercommunalité, je peux vous faire part de l'importance des centres des finances publiques,

Vous me direz certainement que France Services répond à ces besoins, mais nous savons tous, comme cela s'est passé pour les bureaux de poste, qu'il s'agit d'un énième artifice, d'une mesure transitoire vers la mort certaine des services publics dans ces territoires. commission ? Les auteurs de ces trois amendements prévoient de renforcer les crédits du programme 156, 156, relatif à la DGFiP, à hauteur de 160 millions d'euros pour les amendements n II-186 et II-1311, et de 100 millions d'euros pour l'amendement n° II-1350. Le premier motif invoqué est de maintenir les effectifs de la DGFiP, et donc de ne pas supprimer les 1 800 équivalents temps plein prévus pour 2021. Nous y sommes défavorables, pour plusieurs raisons. Le réseau de la DGFiP est engagé dans un profond processus de rationalisation et de réorganisation qui justifie une diminution des effectifs. Cette transformation s'accompagne de la numérisation de certaines démarches-

les effectifs dédiés au contrôle fiscal ont été plutôt préservés ces dernières années, en particulier les emplois les plus qualifiés des directions spécialisées et nationales. Deuxièmement, les moyens déployés dans la lutte contre la fraude fiscale ne sont pas seulement humains, mais aussi technologiques.

ou encore la Mission interministérielle de coordination anti-fraude. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes défavorables à ces amendements. Nous voudrions néanmoins que le Gouvernement apporte des précisions sur la répartition des suppressions de postes prévues en 2021. Pourquoi affectent-elles plus les trésoreries que l'administration centrale monsieur les ministres,

Le parc d'attractions Eurodisney a longtemps été détenu par une société holding immatriculée au Delaware, petit État américain qui compte plus de sociétés enregistrées que d'habitants- ces derniers

Le double effet du renforcement de la contrainte budgétaire à la suite de la crise économique et des gains de productivité qui ont été permis par la dématérialisation n'a pas amélioré la situation. Cela ne veut pas dire que vous avez perdu de l'énergie ou de la volonté. de la volonté. Cependant, le nombre de contrôles sur place est en baisse sensible : « Conséquence de la baisse des effectifs, le nombre de contrôles sur place a connu une forte diminution dans la période récente. Les contrôles sur place des professionnels (vérifications des comptabilités [ ...]) ont baissé de 20 % depuis 2013,

fin du mois. Nous ferons le point plus tard. Votre amendement ne répond pas à un souhait de cette administration. Par ailleurs, s'il s'avérait que les effectifs sont sous-dimensionnés pour répondre au Brexit, les douanes pourraient toujours choisir de recruter ces 100 ETP en 2021, qui ont

que ce soit dans les aéroports ou dans les ports. Du fait de la réduction du volume des échanges, il sera temps, l'année prochaine, de refaire le point. Pour conclure, avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Monsieur le rapporteur

; les crédits de paiement arriveront donc en 2021. C'est le cas pour l'intégralité des projets que nous avons validés en 2019 et 2020. Le décaissement concret des euros sonnants et trébuchants, pour que nous payions des développeurs, pour que nous payions du

je m'attache à ce que nous avancions résolument et que nous livrions en 2022 un État rénové, un État performant, un État qui dépasse les silos ministériels.

le rapporteur pour avis. J'espère que nous partageons tous ici l'idée que l'apprentissage constitue lui aussi une filière d'excellence. Notre pays n'a jamais compté autant d'apprentis : 491 000 contrats d'apprentissage à de 2019, tous secteurs confondus, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Cependant, contrairement aux collectivités territoriales, les ministères ont pris beaucoup de retard en la matière. Il était question en 2016 d'employer 10 000 apprentis. Ce cap n'est toujours pas atteint.

en 2019, en cohérence avec les niveaux de prise en charge déterminés par les branches professionnelles du secteur privé et validés par le nouvel organisme France Compétences. En conséquence, avec cet amendement, nous proposons de recréer la dotation interministérielle qui existait entre 2016 et 2018 elle était alors de 30 millions d'euros ; j'en propose 15 millions -, pour développer l'apprentissage dans la fonction publique de l'État et inciter les ministères à recruter des apprentis en prenant en charge une partie de leur rémunération et de leurs frais de formation. Sur le plan technique, il abonderait

pour intéresser des jeunes à la fonction publique, notamment dans un certain nombre de métiers qui sont un peu sous tension, et pour lesquels il est parfois difficile de recruter. On a parlé à l'instant des projets informatiques : c'est un secteur qui est en forte et l'État a parfois du mal à recruter des informaticiens de bon niveau, parce qu'il y a une forte demande dans le secteur privé et que les concours ne sont pas toujours les plus adaptés. À cet égard, l'apprentissage peut être une solution. Le Sénat lui-même, d'ailleurs, recrute

soutenir notre jeunesse et faire connaître les métiers de la fonction publique, je suis plus que favorable à l'apprentissage. C'est une voie essentielle de recrutement. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les métiers et qui ont une image assez déformée, au fond, de ce qu'est la réalité quotidienne

d'un soutien de 3 000 euros forfaitaires pour tous les contrats d'apprentissage signés entre le 1 juillet 2020 et le 28 février 2021. Avec Élisabeth Borne, je suis très précisément le déploiement effectif, la tuyauterie budgétaire pour que ces crédits soient versés, mais, je tiens à le redire devant vous, ce sont 3 000 euros par apprenti pour tous les contrats d'apprentissage dans la fonction publique territoriale entre le 1 juillet et le 28 février. Votre amendement porte sur les apprentis dans la fonction publique d'État.

des montants pour que les ministères ne soient plus confrontés à une gestion budgétaire extrêmement compliquée, avec des décrets de transfert assez complexes sur la gestion des apprentis.

en tant qu'employeur public. Cela concerne beaucoup de sujets dans mon ministère : la féminisation, sur laquelle je pourrai revenir, la protection sociale complémentaire, un sujet sur lequel je travaille actuellement de manière très résolue avec notamment les organisations syndicales et les employeurs territoriaux, hospitaliers et de l'État. Bref, autant de sujets où nous devons, nous employeurs publics, consacrer les moyens nécessaires pour avoir une fonction publique attractive, mobilisée, et qui prenne sa part dans le recrutement de la jeunesse. Je suis défavorable à votre amendement, parce que je pense que la recentralisation sans les autres mesures autour ne résoudra pas le problème. Nous avons expérimenté le système des décrets de transfert, qui était devenu objectivement extrêmement compliqué. Sachez que je travaillerai vraiment avec vous, madame la rapporteure pour avis, une fois que ce rapport sera remis au Parlement, pour voir ce que nous mettons en oeuvre et m'assurer que le contrôle de l'action du Gouvernement que vous menez est fait avec la plus grande transparence. Madame

Certains vieux bâtiments du parc immobilier de l'État présentent des bilans énergétiques absolument catastrophiques et doivent encore, pour certains, subir des opérations de désamiantage. C'est vraiment d'un autre âge ! Dans le cadre du grand plan d'investissement doté de 1 milliard d'euros, le Gouvernement s'est à accélérer la transition énergétique des cités administratives : une somme de 655 millions d'euros sera, selon l'exécutif, dédiée à la performance énergétique des bâtiments des services publics. Ces travaux permettraient de faire baisser de 50 % les émissions de gaz à effet de serre et de 67 % le montant des factures énergétiques des services.

entraîne souvent la baisse de la qualité du service offert à tous les usagers, surtout pour celles et ceux qui ne peuvent accomplir leur démarche via internet. Cette numérisation des services publics a pour effet pervers d'éloigner les usagers, et nous nous opposons de ce fait à ce choix opéré par le Gouvernement. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande donc que le budget alloué pour la performance énergétique des bâtiments soit spécifiquement dédié à ces travaux de rénovation écologique

nous prévoyons 3,7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique et thermique des bâtiments publics : 950 millions d'euros seront fléchés sur les collectivités dans le cadre d'une procédure qui sera mise en place début 2021 le seront sur les bâtiments d'État et les universités. Bruno Le Maire et moi-même aurons l'occasion, avant Noël, d'annoncer la liste des projets retenus en ce qui concerne l'État, avant la procédure spécifique pour les collectivités. Cela représente plusieurs centaines de projets, puisque tous les projets d'un montant inférieur à 5 millions d'euros ont été décidés à un niveau déconcentré et nous avions reçu 8 000 candidatures, pour un total de 8 milliards d'euros de travaux. Nous en retenons pour 2,7 milliards d'euros, avec un critère

existe bel et bien. Deux décrets prévoient qu'une prime soit attribuée aux agents civils et militaires ultramarins lors de la première affectation en métropole pour les aider à faire face à leurs frais d'installation. Elle est versée à tous les agents ultramarins, sauf ceux originaires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie

Certains renoncent même à s'engager, faute de pouvoir assumer les frais d'installation. Aussi, la ministre de la défense s'est engagée à mettre fin à cette discrimination dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération des militaires, qui sera présentée en 2021, mais elle a besoin de votre concours, dans une approche interministérielle. Gérard Poadja, que je salue, et cosigné par plusieurs élus du Pacifique et par le président de la délégation aux outre-mer, qui est ici présent, nous vous invitons à prendre pleinement part à ce travail pour pour mettre fin à cette discrimination. L'amendement tend à transférer 1 million d'euros d'autorisations d'engagement du programme 352, « Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État », vers le programme 148, qui comprend notamment le fonds en faveur de l'égalité professionnelle créé en 2019.

de ces territoires et pour nous assurer que tous les Français peuvent bien s'engager et servir l'intérêt général, sans distinction. Sur le fond, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont des territoires assez spécifiques,

départements d'outre-mer. D'où cette différence qui a pu exister à l'origine. Le sujet que vous pointez mérite vraiment d'être examiné. Nous devons l'instruire de manière assez précise, notamment pour son chiffrage,

des mesures qui peuvent tout à fait s'entendre, nous abîmions l'attractivité des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie pour les fonctionnaires. C'est aussi important de maintenir des fonctionnaires sur le terrain. Je suis tout à fait favorable à ce que nous travaillions vraiment en détail pour trouver des solutions adaptées, en lien avec les ministères qui recrutent. Je tiens à vous dire que le ministère de la défense a bien identifié la problématique et cherche des solutions dans le cadre de la refonte de la rémunération des militaires. C'est un ministère qui recrute beaucoup en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour faire venir des personnes en métropole ou sur d'autres missions. Je le répète, nous y travaillons. Je pense juste qu'il nous faut

l'on puisse laisser se pérenniser une iniquité flagrante entre ces fonctionnaires, qui servent, j'y insiste, l'État en métropole. Il n'est pas question d'attribuer un budget supplémentaire à la Polynésie française ou aux collectivités du Pacifique. Il n'y a pas de sujet statutaire en l'occurrence. J'ai bien pris note, en tout cas, de la proposition de Mme la ministre de créer un groupe de travail et je suis, bien entendu, volontaire pour y participer, car il me semble qu'en 2021, quand on est fonctionnaire d'État, être né dans le Pacifique ne doit pas être une faute. La parole est

qu'il faut faire des études pour voir si les montants proposés sont suffisants. Lorsque des Wallisiens, qui aiment beaucoup la France et qui s'engagent souvent dans les armées, viennent ici, on ne leur pose pas la question de leur patriotisme. En revanche, ils n'ont pas droit à cette prime. D'ailleurs, madame la ministre, il ne s'agit même pas de prime : il s'agit de traitement indiciaire de base,

est à Mme la ministre. J'entends vos arguments. Je tiens juste à dire, pour que les débats soient éclairés, qu'il n'y a bien sûr aucune différence indiciaire

en préambule. Il vise à réaffirmer, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, l'urgence de suspendre, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les jours de carence dans la fonction publique.

Lors du confinement de mars et avril, et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, le 10 juillet, le Gouvernement avait suspendu cette mesure, mais il a décidé de la remettre en vigueur

le président du Sénat a récemment indiqué, lors d'un déplacement en Haute-Savoie, qu'il était favorable à l'instauration d'une prime de vie chère et à une territorialisation de l'indemnité de résidence. Cette indemnité est régie par le décret du 24 octobre 1985 et la circulaire

est dérisoire, voire indécent : 1 % du traitement indiciaire brut en zone 2, avec un minimum de 14,67 euros ; 3 % en zone 1, avec un minimum de 44 euros. la ministre, que ces montants sont bien loin de compenser les écarts de loyers, notamment pour les jeunes fonctionnaires et tout particulièrement ceux des catégories B et C. La deuxième raison est l'iniquité de cette prime. En effet, certaines régions frontalières ne figurent pas dans le dispositif. Je pense à celle que je connais, le pays de Gex, dans l'Ain, ou aux zones frontalières de Haute-Savoie, qui ne sont classées ni en zone 1 ni en zone 2, alors qu'elles subissent des loyers très élevés du fait de leur proximité avec la Suisse.

que les difficultés d'accès au logement dans le Genevois français aggravent la situation du service public au point de mettre en péril sa continuité dans l'enseignement, la police, le réseau du Trésor public et la santé.

d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale visant à évaluer les conclusions d'un alignement progressif des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles. Le problème est que le rattachement de cet article à la mission « Régimes sociaux et de retraite » est contraire à la Constitution, car il n'entre pas dans le périmètre de cette mission. Malgré l'intérêt majeur de cette question, cet article n'a pas sa place dans une loi de finances ; c'est pourquoi nous vous proposons de le supprimer.

fait prête. Depuis ce vote, qui était très attendu, nous n'avons plus entendu parler de rien.

envisagées pour les recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l'État, correspondant aux retenues sur salaires et aux contributions des employeurs, mais aussi le besoin de financement qui résulterait d'un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés, ou encore les effets qu'aurait le système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes des fonctionnaires. Les textes adoptés par l'Assemblée nationale en mars 2020 sont susceptibles de modifier considérablement la dynamique des recettes et des dépenses des régimes dont le compte d'affectation spéciale « Pensions » retrace les équilibres, ainsi que des obligations et droits qu'entraîne pour les fonctionnaires civils et militaires de l'État leur affiliation à un régime de retraite obligatoire. Ces textes ne sont pas encore définitivement adoptés, mais leur importance est telle, à tous égards, qu'il n'est pas compréhensible que le Parlement puisse demeurer sans visibilité sur les impacts de leur mise en oeuvre sur les dynamiques à long terme des recettes et charges de pension sur lesquelles il est appelé à exprimer son vote.

la réforme des retraites a été suspendue. Il nous paraît extrêmement compliqué de produire des informations sur un texte qui ne fait pas l'objet d'un examen parlementaire, même s'il avait fait l'objet d'une étude d'impact volumineuse qui abordait largement les sujets que vous évoquez.

J'entends bien la réponse que nous fait M. le ministre, mais je m'étonne quand même qu'il puisse refuser des éléments d'information au Parlement. Soulignons que le Conseil d'État lui-même s'était étonné du

l'article 74. Tous les crédits afférents aux missions ayant été examinés, le Sénat va maintenant statuer, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, sur les articles qui portent récapitulation de ces crédits. Je vais appeler les articles 33 à 36 et les états B à E qui leur sont respectivement annexés, relatifs aux crédits et découverts pour 2021. La direction de la séance du Sénat a procédé à la rectification des états B et D, de manière à tenir compte des votes qui sont intervenus lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances.

Je voulais profiter de son examen, monsieur le ministre, pour vous faire part de ma préoccupation concernant certains opérateurs à qui vous demandez de faire plus et, parfois, beaucoup plus dans le cadre de la relance, tout en baissant leur plafond d'emplois,

Certes, dans le cadre du plan Action publique 2022, il était prévu que VNF diminue ses effectifs d'une centaine d'ETP par an,

assignés à cet opérateur peuvent à première vue apparaître relativement réalistes. Je note toutefois que la diminution prévue en 2021 est particulièrement forte, ce qui suscite des inquiétudes légitimes chez VNF, car beaucoup d'installations nécessitent des interventions humaines. En outre, élément important, VNF va voir son niveau d'investissement considérablement augmenter en 2021 et en 2022 dans le cadre du plan de relance, puisque celui-ci devrait permettre la réalisation de quelque 160 projets sur le réseau géré par cet établissement.

nous ne souhaitons pas que la mise en oeuvre du plan de relance se traduise par des recrutements pérennes qui viendraient sédimenter, pour la suite, de la dépense publique sous forme de masse salariale.

Tout comme l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), qui réclame aujourd'hui plus de moyens, l'Agence Bio est sous-financée. Un rapport d'information du Sénat remis en janvier dernier sur les financements de l'agriculture biologique avait d'ailleurs bien noté, pour l'ITAB comme pour l'Agence Bio, un déficit récurrent des moyens disponibles pour accomplir leurs missions, le changement d'échelle de la production biologique et des besoins de pilotage subséquents insuffisamment pris

effet, peut-il être proposé de donner moins de moyens à la Société du Grand Paris, alors même que la commission des finances a rendu récemment un rapport rappelant l'importance et l'urgence d'attribuer des moyens et de structurer cet établissement ?

Devant nous, des problèmes vont s'accumuler, notamment sur la pollution, qui est en train de croître. Force est de constater que des communes et des syndicats